La parole est à Mme Nathalie Goulet,

y le ZAN, et l’on aboutit à des situations inextricables. Mes chers collègues, soyons responsables, nous aussi : assumons les conséquences de la disparition de la taxe d’habitation et de la mise en œuvre du ZAN, et laissons les communes décider librement de leurs taux et de leurs impôts

Monsieur le ministre,

n° I 503 rectifié . Dans la même lignée, cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants

neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation ou encore simplifier le travail des services fiscaux de l’État et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités. Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, incitent soit à l’artificialisation, soit à l’étalement urbain. Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

sur les logements vacants abondant aujourd’hui le budget général de l’État, il est enfin proposé que les collectivités territoriales compensent l’État pour la perte du produit de la TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.

l’un des seuls domaines dans lequel les exécutifs locaux exercent encore des responsabilités. Cet amendement tend ainsi à fusionner la taxe sur les logements vacants, qui concerne aujourd’hui exclusivement les communes de plus de 50 000 habitants listées par décret, et la taxe d’habitation sur les logements vacants, qui peut être instaurée dans toutes les communes où la la taxe sur les logements vacants n’est pas appliquée. La TLV vise les communes marquées par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Or ce critère est flou. Il crée de l’insécurité pour les élus locaux, même si une part importante des communes éligibles ont instauré La modification de zonage intervenue l’année dernière permet un élargissement bienvenu à près de 2 000 communes supplémentaires.

peut être un outil d’indexation du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite

qui sont soumises à la crise du logement la plus dure : dans les zones littorales, à Paris, dont je suis l’élu, dans un certain nombre de communes touristiques, notamment dans les Alpes, sur la Côte d’Azur, sur le littoral atlantique.

ajoutée des entreprises (CVAE), non pas parce que les élus locaux auraient une appétence pour les taxes, mais parce que nous avons une appétence pour l’autonomie fiscale,

que des zones entières du territoire soient tellement sujettes au développement des résidences secondaires, à « l’airbnbisation », en raison de leur attractivité touristique et économique, que les gens n’arrivent plus à s’y loger.

des départements pour lesquels les ressources fiscales sont vraiment devenues marginales, c’est bien parce que nous voulons que les conseils municipaux puissent moduler les taux. Cet amendement vise à leur permettre de le faire pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans pour autant augmenter nécessairement la taxe sur le foncier bâti, qui touche aussi bien les propriétaires de maisons d’habitation que les artisans et les entreprises. le faire dans une certaine limite, car nous sommes des gens raisonnables. Nous ne voudrions pas que les taux doublent pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. C’est pourquoi nous proposons que la liberté existe

d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans toucher à la taxe foncière. Monsieur le ministre, je vous remercie de ne pas faire notre procès et vous m’excuserez si je fais un peu le vôtre. Le lien fiscal est un lien démocratique. Si votre idéal est d’assujettir le financement des communes, des départements, des régions à des décisions de l’État, nous ne le partageons pas. Nous considérons que la suppression de la taxe d’habitation est une erreur historique. Nous considérons que, lorsque nos habitants ont besoin de nouveaux équipements et services, ils ont à les payer. Nous considérons que les équipes municipales mettent

sur les résidences secondaires. Eh bien, monsieur le ministre, oui, nous avons une profonde divergence de vues sur la question de la confiance à accorder aux élus municipaux et à la démocratie locale.

lorsqu’à la suite d’une fusion d’intercommunalités le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences secondaires était supérieur en 2020 de plus d’une franchise de 2 % au taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette distorsion était de nature à occasionner une perte pérenne de ressources fiscales aux intercommunalités issues d’une fusion antérieure à 2019 et pour lesquelles la taxe d’habitation sur les résidences principales avait été indemnisée par une fraction de TVA sur la base d’un taux moyen pondéré très inférieur au taux moyen pondéré résultant de la prise en compte de l’ensemble des bases de taxe d’habitation existant en 2020. L’amendement qui vous est proposé vise à corriger le désagrément induit par la réforme pour les EPCI qui sont dans cette situation et ajuster les impacts de la réforme le temps du lissage des taux. Il permet aussi de réaffirmer l’objectif de neutralité sur les recettes des collectivités locales de la réforme de la taxe d’habitation, qui n’est pas assurée. L’effort financier ne repose pas sur le budget de l’État de réajuster la contribution des contribuables à la hauteur du lissage des taux, de régler de manière structurelle la fragilité des ressources des EPCI et d’écarter tout risque contentieux.

des inégalités extrêmes de notre société : aujourd’hui, des gens travaillent, mais ne peuvent plus accéder à la propriété, alors que d’autres peuvent